La séance est reprise. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Adrien Giraud, qui fut sénateur de Mayotte de 2004 à 2011. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire. Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 1 A.

Au moment où le Gouvernement a annoncé la reprise de 35 milliards d'euros de la dette au cours du quinquennat, il convient de s'assurer que cette dette ne puisse pas se reconstituer.

de 2017, la dette de SNCF Réseau avait dépassé 46 milliards d'euros. Cette augmentation continue s'est accélérée depuis 2010,

Le sujet de la dette a été identifié très tôt puisque, dès 1991, un service annexe d'amortissement de la dette ferroviaire était créé.

Cette mesure de protection a été renforcée en 2014 par l'inscription dans la loi d'une « règle d'or ». Elle précise que, tant que la dette de SNCF Réseau dépasse un certain plafond, SNCF Réseau ne peut contribuer au financement des projets de développement, qui doivent donc être financés par l'État et les collectivités. Tout cela n'a pas suffi.

termes, alors que, depuis dix ans, le montant de la régénération du réseau a triplé, passant de 1 à 3 milliards d'euros par an, ce qui était indispensable, les ressources de SNCF Réseau n'ont pas suivi. C'est à ce décalage qu'il faut remédier. Nous le faisons, d'une part, en reprenant

son retour à l'équilibre, qui sera maintenu sur la durée. Cette trajectoire de retour à l'équilibre, qui permet de financer le programme d'investissements de SNCF Réseau, sera, bien sûr, inscrite dans le nouveau contrat de performance entre l'État et cet

Ce qui est évident dans le débat qui nous intéresse, c'est, bien sûr, que le mouvement des cheminots peut toujours s'essouffler, à en croire les informations officielles, mais qu'il aura eu comme résultat, entre autres, d'amener le Gouvernement à se pencher sur la dette du groupe SNCF et, singulièrement, celle de SNCF Réseau ! Le montant de la dette d'infrastructures est connu : 46,6 milliards d'euros, soit l'équivalent de 2 points de PIB aujourd'hui, que SNCF Réseau a incontestablement porté depuis 1982, en lieu et place de l'État. En effet, la dette des entreprises publiques, qu'il s'agisse de celle d'EDF, de la SNCF ou de toute autre du même type, provient, de manière quasi exclusive, de la clause d'autonomie de gestion qui leur a été imposée, dans un contexte de forte inflation et de dérégulation des marchés financiers, ce qui ne retire rien au fait que la gestion de la dette de SNCF Réseau a été globalement menée avec un professionnalisme certain. À tel point, mes chers collègues, et c'est peu connu, qu'elle est en partie constituée d'obligations de très longue durée et que sa durée de vie moyenne s'avère plus importante que celle de la dette de l'État. Le rapport remis en août 2016, en application de l'article 11 de la réforme ferroviaire d'août 2014, montre que SNCF Réseau n'a pas grand bénéfice à tirer d'une simple reprise de sa dette par l'État, l'État, qu'il s'agisse de la durée de vie de la dette, mais aussi du taux d'intérêt qui la grève et des outils de refinancement mobilisés pour sa gestion active. La signature de SNCF Réseau est de bonne qualité sur les marchés financiers, d'autant que les trois quarts de l'encours de la dette sont libellés en euros, ce qui n'expose donc l'établissement public qu'à un risque de charge quand même limité. Autant dire que la solution choisie par le Gouvernement a tous les défauts de l'exercice obligé. En effet, nul ne l'ignore désormais, le toilettage des comptes, notamment du bilan de la SNCF Réseau, est étroitement lié au changement de nature juridique. De plus, la fameuse règle d'or risquerait de venir s'appliquer, anéantissant toute possibilité d'emprunt sur le court et moyen terme. Nous proposons une solution avec cet amendement. J'espère qu'il retiendra votre attention, monsieur le rapporteur, madame la ministre.

le taux de retour sur l'investissement pour SNCF Réseau doit être « au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l'investissement

Dans un cas, SNCF Réseau continue de participer à la solidarité nationale territoriale. Dans l'autre, elle se trouve extrêmement encadrée et seuls l'État et les collectivités territoriales

subsister au bilan d'entrée de SNCF Réseau une dette proche de l'amener à des fonds propres nuls et, surtout, vous ne touchez pas à la dette de SNCF Mobilités, dont on sent confusément qu'elle va être amortie par le dépeçage du réseau secondaire- entre autres -et des équipements roulants y afférents que le présent texte de loi organise. Nous sommes, pour notre part, partisans d'une association précise entre l'expertise du service financier de SNCF Réseau et l'expérience et les références des cadres, techniciens et agents de la Caisse des dépôts et consignations. Vous le voyez, madame la ministre, nous ne sommes pas seulement dans une attitude d'opposition. Nous vous soumettons des propositions alternatives. À cette association, donc, de faire en sorte que le financement des opérations d'investissement de SNCF Réseau soit bouclé dans les meilleures conditions et que le refinancement de la dette en découlant puisse notamment être mis en oeuvre auprès de la Banque centrale européenne. Celle-ci, ne l'oublions pas, a mis en oeuvre, depuis plusieurs années, un dispositif de création monétaire appelé, qui a qui a pourvu les acteurs bancaires et financiers de rien moins que 2 486 milliards d'euros, soit bien plus, pour ne donner qu'un exemple, que la dette publique de notre pays, tous émetteurs confondus ! Cette opération s'est soldée, entre autres, pour la BCE, par l'acquisition, sur le second marché, de titres de créances publiques et privées. Il n'est même pas interdit de penser que les opérations de la Banque de Francfort n'aient amené à acquérir des titres de dette publique française, de celle d'EDF ou encore de la SNCF, en la rendant de fait plus « soutenable ». Soyons précis ! La BCE se tient aujourd'hui sur un taux directeur fixé à zéro, prend en charge les disponibilités bancaires avec un taux négatif de trente à quarante points de base, et est en situation de pouvoir travailler avec la Caisse des dépôts Elle pourrait d'ailleurs, pour le coup, déployer une action plus large sur l'ensemble des opérateurs du secteur ferroviaire en Europe. Voici exposées un certain nombre de raisons qui font que nous sommes en désaccord, madame la ministre, avec ce que vous proposez dans votre amendement et, en même temps, nous ne sommes pas seulement contre votre réforme, nous sommes pour une autre construction.

vote. Je tiens à le redire, le désendettement est possible. Il est lié à l'amélioration de la situation du déficit public. Il est important, dans ce moment précis du débat, de le rappeler. Je tiens aussi à saluer les propos de M. le rapporteur sur l'origine de la dette, car je les partage totalement. J'ai plusieurs questions à poser. Tout d'abord, vous améliorez la règle d'or mise en place en 2014.

Qu'en est-il de la trajectoire financière de SNCF Mobilités, qui n'est pas allégée ? Les 35 milliards concernent SNCF Réseau. Qu'en est-il de sa future trajectoire financière ? Nous demandons des engagements précis à ce niveau. Puisqu'on parle de soutenabilité de la dette, j'ai besoin de comprendre la démonstration arithmétique au terme de laquelle cette reprise

Or la dette, selon la trajectoire financière établie dans le contrat de performance signée avec l'État, sera à un niveau de près de 10 milliards d'euros supplémentaires. Il restera donc à charge pour l'entreprise non pas 15 milliards mais près de 25 milliards d'euros. Cela, si j'ose dire, relève d'un autre débat ... Le pendant de cette annonce, c'est cet amendement qui modifie la fameuse règle d'or décidée en 2014 par un décret paru en mars 2017 qui conditionnait les possibilités d'investissement à un ratio entre l'endettement net de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle. Ce nouvel amendement prévoit de limiter davantage les capacités d'investissement en se fondant sur la couverture du coût moyen pondéré du capital- en clair, du taux de profitabilité de l'investissement : un euro investi doit rapporter au moins un euro. C'est la confirmation de la mise à mort des lignes ferroviaires de proximité de nos territoires : on renvoie leur financement aux seules collectivités territoriales, qui sont déjà, vous le savez, mes chers collègues,

Nous proposons, pour notre part, une autre stratégie pour SNCF Réseau. En effet, son désendettement ne créera pas d'appel d'air pour financer la nécessaire rénovation et régénération des lignes. Comme nous ne faisons pas que nous opposer

D'abord, je répondrai à Ronan Dantec et aux autres orateurs qui semblent considérer que c'est à SNCF Réseau de prendre en charge l'aménagement du territoire. Non !

pèse sur les gouvernements successifs qui ont laissé à SNCF Réseau ou, auparavant, à Réseau ferré de France le soin de prendre en charge des missions d'aménagement du territoire, ce qui n'était pas leur rôle. Sur la question de la dette, je voudrais à mon tour saluer l'effort fait par le Gouvernement

oui, il faut une règle d'or, oui, il faut que nous la votions, mais il faut aussi que le Gouvernement mette ensuite tout en oeuvre pour qu'elle soit respectée et appliquée pleinement. En effet, c'est très bien de reprendre la dette, mais il faut surtout éviter qu'elle ne se reconstitue, sans quoi, dans dix ans, on en sera au même point. La parole est à Mme la ministre.

J'ai bien entendu vos exposés sur la complexité des produits financiers en Europe. Pour ma part, j'en retiens cela : finalement, vous ne souhaitez pas avoir de débat, et vous êtes incapables d'admettre qu'il y a au moins un point sur lequel nous pouvons être d'accord, savoir la volonté du Gouvernement de soulager le système ferroviaire d'une partie très substantielle de sa dette pour lui donner la capacité d'investir davantage et de se développer. Même sur ce point-là, vous ne pouvez pas être d'accord avec nous ! Personne n'a dit cela ! Votre amendement vise

du secteur ferroviaire : nous comptons sur une amélioration de la performance et une réduction de l'écart de compétitivité entre la SNCF et ses homologues. Le Premier ministre a mentionné

sur l'article. Aujourd'hui, le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel régit les conditions d'embauche, de rémunération et de déroulement des carrières, les sanctions et garanties disciplinaires, la mobilité géographique et fonctionnelle inhérente à l'entreprise nationale, les congés, les conditions de cessation de fonction, l'assurance maladie et le droit syndical. Le statut donne des droits, mais il confère aussi des devoirs : la période d'essai est d'un an, et même de trois ans pour les cadres ; le travail du dimanche et des jours fériés est rémunéré en dessous du code du travail. Ajoutons le travail de nuit et la mobilité induite. Aujourd'hui, la grille de rémunération place environ 3 000 cheminots à un niveau inférieur au SMIC

les cheminots sont soumis sont atypiques ; en outre, ils ont l'obligation de faire fonctionner la SNCF toute l'année. Si la sécurité ferroviaire et la continuité du service sont les fondements du statut des cheminots de la SNCF, il faut y ajouter un principe de neutralité. En effet, les cheminots ne travaillent pas, en principe, pour répondre à des exigences patronales ou financières ; ils s'engagent pour placer l'entreprise publique au service de la Nation et des citoyens. Cela suppose que l'agent de la SNCF reste en responsabilité et ne soit pas soumis à des aléas relevant de l'arbitraire technocratique ou financier. chers collègues, mettre un terme à cette logique de fonctionnement et d'investissement professionnel ?

à son « effort de redressement » et une contrepartie à la reprise de la dette ferroviaire annoncée par le Premier ministre lui-même. L'économie réalisable s'établirait entre 10 et 15 millions d'euros par an : sur la durée moyenne de vie de la dette de SNCF Réseau,

sur le réseau de l'État et fut généralisé en 1920 à l'ensemble des compagnies. Il est donc bien antérieur à la création de la SNCF. Il faut le distinguer du régime spécial des retraites des cheminots, dont l'origine remonte à 1909, qui ne lui est pas directement lié, bien qu'il assimilé. Le statut s'apparente davantage, dans sa forme, à une convention collective dont la spécificité est de relever d'un acte réglementaire gouvernemental. Ces règles ont été maintenues lors de la nationalisation de la SNCF.

nécessaire un statut national, qui répondait également au besoin d'établir des règles unifiées dans un secteur essentiel à la marche globale de l'économie du pays et à son aménagement territorial. Cela Cela a conduit l'État à légiférer pour créer un statut unique à l'ensemble des travailleurs du ferroviaire. Il a ainsi imposé aux différentes compagnies d'employer un nombre d'agents suffisant de les fidéliser pour permettre la transmission des savoirs et savoir-faire professionnels. Chaque cheminot doit ainsi avoir un haut niveau de formation, au regard des spécificités fortes des différents métiers, et l'organisation du travail doit être encadrée afin de garantir la sécurité

Roland Courteau, qui ne peut être présent à cet instant et qui souhaitait lui aussi vous faire part de son opinion sur la proposition qui nous est faite. Pourquoi le Gouvernement veut-il imposer à la SNCF cette réforme doctrinaire qui met à terre tant le statut de l'entreprise que celui des cheminots ? Pourquoi diable ce gouvernement veut-il être celui qui aura eu la tête du mythique statut des cheminots et du service public à la française ? On nous dit que c'est l'Union européenne qui le veut. l'Union européenne qui le veut. Une fois encore, elle a bon dos ! Ni la réforme du statut des cheminots ni la transformation de la SNCF en société anonyme ne sont nécessaires. Dès lors, et comme cela a été dit, j'aurais tendance à contester le texte, le contexte et, surtout, le prétexte ! Que des évolutions soient nécessaires, cela peut s'entendre, mais elles ne doivent pas être conduites n'importe comment et à n'importe quel prix. Or le prix, à ce jour, est énorme ! On peut, comme l'a dit mon collègue Olivier Jacquin, dynamiser la SNCF sans la dynamiter ! Ce que l'on peut reprocher aux auteurs de ce texte, c'est de vouloir tirer argument de l'ouverture à la concurrence pour modifier le statut, alors qu'il n'y a aucun lien à établir. Vous ne pouvez pas prétendre que le statut des cheminots est à l'origine des difficultés financières de la SNCF. Nous sommes nombreux ici à le contester. Saluons plutôt les cheminots, qui servent la SNCF et font que les Français aiment le train Ces hommes du rail ne sont pas des privilégiés, mais l'avant-garde d'un mouvement de préservation des biens communs et de l'intérêt général. Dois-je rappeler, par ailleurs, que le gouvernement précédent s'était engagé, en 2014, à construire un cadre social commun et homogène à l'ensemble du secteur ferroviaire, avec maintien du statut des cheminots ? Que ne l'a-t-il fait ? ... Oui, nous contestons et le texte, et le prétexte ; l'Union européenne ne demande pas

que le statut de cheminot fait partie de notre imaginaire collectif et que c'est un bien commun de la société française. Cela ne signifie

SNCF Réseau et SNCF Mobilités n'auraient pas actuellement des difficultés de recrutement. Il faut savoir que, comme cela a été rappelé, les salaires de début de carrière sont tellement faibles que, pour certains métiers de la SNCF, on a aujourd'hui du mal à recruter,

comme cela a été le cas pour le transport routier avec les dispositifs de cabotage, doublés par le recours aux travailleurs détachés. Nous sommes donc favorables à une évolution,

Nous sommes dans une situation de conflit grave, et il ne faut pas s'en étonner. Imaginez-vous vivre, dans vos professions et métiers respectifs, le climat d'incertitude dans lequel on a placé les cheminots ? Je suis agriculteur. Imaginez que, demain, la coopérative à laquelle je livre des céréales- pas assez cher

vous sera présentée dans quelques minutes : nous entendons conditionner la fin du recrutement au statut à la signature effective d'une convention collective ferroviaire négociée. Nous proposerons un certain nombre d'amendements de repli. Réfléchissez : c'est pragmatique, j'en ferai la démonstration.

sont financés par les cheminots et les cheminotes eux-mêmes. Il n'y a donc pas, là non plus, matière à casser leur statut. Enfin, je ne sais pas ce qu'on leur reproche

On a entendu beaucoup de choses sur le statut des agents. L'étude d'impact estime qu'il occasionnerait des coûts élevés que n'auraient pas à supporter des entreprises concurrentes qui recruteraient des agents

qui dépassait les limites, on peut comprendre que cette profession a réagi et est actuellement dans la rue. Nous nous opposons

quelques vérités. La logique des choses, c'est la suppression du recrutement au statut, mais le statut ne va pas disparaître.

Jacquin, il faut éviter de créer de la confusion. Or vos propos laissaient entendre que nous étions en train de remettre en cause le statut des cheminots qui travaillent aujourd'hui à la SNCF. Il n'en est pas question

Vous pouvez être contre, mais vous allez bientôt voter l'ouverture à la concurrence du secteur. Cela signifie que, dans ce secteur, se trouveront d'autres entreprises qui auront des salariés exerçant les mêmes métiers et ayant par conséquent les mêmes contraintes.

avant la fin de l'année 2019, une convention collective de haut niveau qui s'applique de façon équitable à l'ensemble des salariés de la branche. Par conséquent, il émet un avis défavorable sur ces amendements

En aucun cas, le statut de la fonction publique n'est remis en question, mais nous constatons partout, dans tous les ministères, qu'aujourd'hui les agents qui travaillent dans le service public et qui sont embauchés ne le sont plus sous statut de la fonction publique. On en arrive à un niveau de précarisation que même le privé ne connaît pas ! S'agissant de

ma collègue Laurence Cohen : ce sont deux visions de la société qui s'affrontent. Vous voyez, madame la ministre, on vous écoute, on vous comprend, mais on ne partage pas.

de décembre 2019 il n'y aurait plus de recrutement au statut. Or, selon le projet de loi que nous sommes en train de voter, les transferts de SNCF Mobilités à de nouveaux opérateurs

sauvage, mondialisée, liée notamment au travail détaché et au cabotage. Nous sommes dans un secteur non délocalisable par définition et non soumis à la concurrence mondiale. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de dumping social dans ce domaine.

je rejoins ce qui vient d'être dit : on ne peut pas prendre comme argument le principe d'équité quand on s'apprête à mettre en place au sein d'une entreprise une situation où l'équité et l'égalité entre les salariés auront disparu, et ce pour de nombreuses années

que ceux-ci ont le statut de fonctionnaire ou relèvent de la convention collective. Il ne vous a pas échappé que, dans les amendements qui ont été introduits en commission, j'ai souhaité promouvoir ces principes d'unité sociale auxquels les syndicats qui ont bien voulu être dans une position de dialogue sont attentifs. Par conséquent, il y aura bien, au sein de la SNCF, un socle de droits communs et des modalités différentes selon que l'on est au statut ou que l'on dépend de la convention collective, avec des équilibres qui peuvent être différents.

repli, qui vise à garantir qu'il n'y ait pas de perte de droits et qu'il ne soit pas mis fin au statut des cheminots pour les nouveaux personnels tant qu'une règle commune de branche n'a pas été négociée à droits équivalents. Par conséquent, la référence au 31 décembre 2019

Aussi bien les organisations syndicales que les organisations patronales considèrent qu'il sera difficile d'aboutir dans des délais aussi serrés à la conclusion des accords collectifs au regard des négociations actuelles. La date de 2019 n'étant donc pas réaliste, nous proposons un délai plus raisonnable, permettant de prolonger les négociations jusqu'au 31 décembre 2023. Qui plus est, la période entre 2019 et 2023 constituant dans une certaine mesure une période expérimentale de l'ouverture à la concurrence en raison de sa progressivité et de ses spécificités géographiques, que les négociations puissent se prolonger durant cette période pour assurer la réussite des accords collectifs qui permettront d'éviter le dumping social, en assurant les garanties sociales pour l'ensemble du personnel de la branche ferroviaire. Nous souhaitons donc conditionner la date d'extinction du recrutement

est, certes, un peu court, mais réalisable, car nous ne partons pas de rien : la négociation de cette convention collective a démarré en 2014 et quatre accords ont d'ores et déjà été conclus et étendus par arrêté ministériel, en particulier des accords relatifs à l'organisation du travail et à la formation professionnelle. Les autres volets sur lesquels la négociation devra aboutir concernent notamment les classifications et rémunérations, les garanties collectives des salariés de la branche et le droit syndical.

entendu un représentant du syndicat des patrons du ferroviaire, l'UTP, me dire à peu près la même chose et me confier qu'il ne comprenait pas

tel transfert. C'est là-dessus que la discussion bute, achoppe, ce qui crée ce climat d'incertitude extrêmement fort. C'est pour cette raison que nous proposons ce premier amendement de repli, pour donner une chance à la négociation et, surtout, arrêter le conflit.

Nous allons au bout de notre idée, mes chers collègues, en présentant un ultime amendement de repli pour proposer une date limite de fin de négociation qui corresponde aux pratiques

il ne me paraît pas sérieux, alors que la négociation est engagée depuis 2015, que la discussion a déjà eu lieu sur les classifications et les rémunérations, et que des

Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote. Je voudrais renchérir sur ce que vient de dire mon ami Claude Bérit-Débat. Madame la ministre, le Sénat a toujours eu la réputation de trouver le point d'équilibre entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. De notre avis,

et j'inclus les syndicats des entrepreneurs. Il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance aux partenaires sociaux et de ne pas leur donner le temps nécessaire pour aboutir à un accord raisonnable et équilibré. Je mets

Le scrutin est ouvert.

en cours de négociation, pour tenir compte de la transformation du groupe public ferroviaire prévue à l'article 1 A. Par ailleurs, il étend l'application du décret-socle et de la convention collective aux entreprises dont l'activité principale est est la maintenance des matériels roulants, hors réparation, ou l'exercice de fonctions de sécurité ferroviaire. Quoi qu'il en soit, nous refusons absolument le changement de statut de l'entreprise publique, considérant que ce statut d'EPIC est lié à la nature même de son activité, un service public répondant à l'intérêt général. Plus particulièrement, il s'agit du service public de mobilité, qui est aussi un droit pour nos concitoyens. Nous proposons donc, en cohérence avec l'ensemble de nos amendements, la suppression de cet article, pour pouvoir attendre l'issue des négociations avec les syndicats.

de statut ! Cela passe par un changement de statut, puisque la réforme précédente a bien démontré l'impossibilité d'avoir une unité au travers de trois EPIC. Je voudrais attirer votre attention sur l'importance de l'article que vous voulez supprimer, puisqu'il s'agit d'adapter le champ du décret-socle

Cela se justifie, d'une part, du fait des passifs des différentes privatisations et ouvertures à la concurrence dans le secteur de l'énergie, des communications ou même du fret ferroviaire. Comment oublier, par exemple, la récurrence des suicides sur le lieu de travail constatée dans les années suivant le recul de l'État à France Télécom ? Ces drames humains doivent nous rappeler que, lorsque l'État se retire d'un secteur économique, c'est tout un modèle qui change et des vies qui, parfois, tanguent. Cela est nécessaire, d'autre part, car les expériences étrangères démontrent une détérioration du service et des conditions de travail. La libérale liant la concurrence à une meilleure sécurité et des prix plus intéressants, si elle se fonde sur des principes économiques hérités d'Adam Smith, oublie un détail important. Le secteur privé vise le profit et uniquement le profit. Cela implique donc la recherche absolue de la rentabilité, comme l'ont montré les exemples britannique et allemand hausse des tarifs, investissements moindres sur des lignes jugées peu rentables, problèmes de sécurité, dysfonctionnements répétés. On ne peut nier qu'aujourd'hui 60 % des Britanniques souhaitent une renationalisation du réseau. L'image d'une SNCF toujours en retard, dépassée, honnie et pratiquant des tarifs prohibitifs est à interroger. Oui, au fil des années, le désengagement de l'État et les choix stratégiques faits par ses cadres, dont un certain nombre sont d'ailleurs au Gouvernement aujourd'hui, ont détérioré le service. Malgré toutes ces difficultés, la SNCF reste un bel outil, comme l'a montré dans un rapport le Boston Consulting Group, qu'on ne saurait qualifier de gauchiste. En classant le réseau français troisième réseau le plus performant d'Europe derrière ceux de la Suisse et de la Suède, il a rappelé que la qualité et la sécurité ce réseau étaient dues à l'investissement public et général, et au monopole d'État. Une qualité de service, certes, chancelante, mais supérieure à celle de ses voisins, des exemples peu rassurants de l'étranger, l'enjeu de l'ouverture à la concurrence est central dans nos débats. Dans ce cadre, nos positions doivent s'appuyer sur des études complètes, que seuls nos partenaires européens peuvent nous fournir. Pour cette raison, nous demandons la réalisation d'un bilan contradictoire de ces politiques de libéralisation. Quel est l'avis de la commission ? Mes chers

vous l'indiquer. Sur le fond, plusieurs bilans ont déjà été effectués sur l'ouverture à la concurrence. Ils ont relevé ses effets positifs sur la qualité du service rendu ou la réduction des coûts, au profit des usagers.

en face et préparer l'entreprise et les salariés afin que cette ouverture à la concurrence soit une réussite pour les voyageurs, les territoires, la SNCF et les cheminots.

que ce transfert d'actifs vers l'État soit la contrepartie de la reprise de la dette à hauteur de 35 milliards d'euros, mais, dès lors, comment sécuriser juridiquement la relation entre un État propriétaire

modifier les missions, l'organisation, la forme juridique et la gouvernance de la SNCF. Nous discutons de toute une série de questions très importantes, mais, au final, on nous demande d'emblée, dans l'article 1du texte,

Il a finalement opté pour une méthode inédite consistant à réintégrer certaines dispositions initialement prévues dans le champ de l'ordonnance. Le projet de loi, dont le volume a quasiment quadruplé, est devenu un texte hybride, hétérodoxe, entre articles portant habilitation à légiférer par ordonnance et articles classiques, ce qui n'améliore pas la clarté du texte. Le champ des ordonnances continue d'augmenter au fur et à mesure que de nouveaux articles viennent gonfler le projet de loi. Opposés aux ordonnances, nous considérons que le Parlement doit pouvoir jouer pleinement son rôle sur une réforme ferroviaire aussi importante que celle de la transformation de l'organisation du groupe et du régime juridique des personnels. C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article. Le débat parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, a fait considérablement

du Gouvernement ? On peut raconter l'histoire à l'envers et laisser penser qu'on a ajouté des ordonnances au fur et à mesure du débat parlementaire. En réalité, c'est tout le contraire. Dès le départ, le Gouvernement avait indiqué

souhaitions remplacer les habilitations à prendre des ordonnances par des articles de loi. C'est ce qui s'est produit tout au long du processus parlementaire, d'abord à l'Assemblée nationale, puis en commission au Sénat. Ainsi que M. le rapporteur vient de le souligner,

Le scrutin est ouvert.

Lors des débats sur la loi ferroviaire du 4 août 2014, pour ne reprendre que la législation la plus récente, la nécessité d'un groupe ferroviaire unifié a enfin été reconnue. dix-sept années d'éclatement de notre système ferroviaire, un constat s'est imposé : le démembrement du service public a entraîné une dégradation sans précédent du réseau, des fermetures de ligne et une baisse certaine de la qualité de service. Le cloisonnement des métiers et des personnels ainsi que le recours massif à la sous-traitance d'activités essentielles ont mis à mal la complémentarité des métiers et des savoirs, ce qui a abouti à des inquiétudes, des souffrances et des dysfonctionnements. Pour notre part, dans une démarche constante et cohérente, nous n'avons jamais cessé de pointer les lacunes de la réforme de 1997 : poids des intérêts divergents de RFF et de la SNCF, perte d'énergie dans la gestion des relations entre deux entreprises publiques, qui devaient logiquement travailler ensemble, et remise en cause de la légitimité des cheminots. La séparation en trois EPIC, qui annonçait l'éclatement de la SNCF et sa privatisation, loin de l'objectif d'amélioration du système ferroviaire, a seulement multiplié les structures de coordination, d'arbitrage ou de consultation. Comme cela a été largement souligné, la gestion par activité n'est pas pertinente dans un système ferroviaire mixte, où les trains de toute nature empruntent les mêmes voies, où les locomotives et les conducteurs peuvent tracter tout type de matériel roulant et au sein duquel l'exploitation ferroviaire est assurée par les agents de la même filière, quels que soient les trains. En bref, il ne s'agissait à l'époque que de préparer la vente à la découpe du rail français. En effet, la privatisation des services publics en réseau a été systématiquement accompagnée du démantèlement de l'opérateur historique en plusieurs entités. Nous pensons que l'intégration étroite et réelle est la seule voie raisonnable et pragmatique, ni idéologique ni régressive, pour assurer l'efficacité indispensable de ce grand service public qu'est le chemin de fer français. C'est pourquoi une nouvelle réforme de l'entreprise historique ne doit avoir pour seul objectif que de mettre fin à une organisation qui a déjà démontré son inefficacité. Le service public que nous défendons englobe non seulement l'offre de services, la gestion et le déploiement des réseaux,

M. Fabien Gay. Le 28 février dernier, le CESE a rendu un avis alarmant sur l'application de la loi relative à la transition énergétique votée en 2015. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici à 2030 et de 75 % à l'horizon de 2050 seront inatteignables en l'absence d'investissements majeurs, notamment dans les alternatives aux transports routiers individuels. Le présent projet de loi s'inscrit dans un mouvement inverse, alors que nous savons que notre réseau ferroviaire est un atout majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique- nous l'avons dit tout à l'heure -et, plus localement, pour la qualité de l'air dans nos métropoles. C'est également ce qu'expliquent, dans une tribune au, Pascal da Costa et Elwyn Sirieys, respectivement enseignant-chercheur et élève ingénieur à CentraleSupélec- peut-être leur accorderez-vous un crédit légèrement supérieur à celui que vous accordez aux syndicats ou aux parlementaires que nous sommes ... De toutes les critiques adressées au projet de réforme, le respect de l'environnement est celle dont on parle sans doute le moins. Or, comme Or, comme l'étayent ces deux scientifiques, alors que le réseau ferroviaire représente aujourd'hui près de 10 % du volume de transport sur le territoire métropolitain, il n'est à l'origine que de 0,52 % du CO2 imputable aux transports et de 6 % des émissions de particules fines de type PM10. Le refus du Gouvernement de reprendre à son compte des objectifs du Grenelle de l'environnement, qui proposait de faire passer la part modale du non-routier et du non-aérien de 14 % à 25 % d'ici à 2022, et la volonté affichée de restreindre le domaine de pertinence du ferroviaire à partir de considérations financières et comptables emportent des conséquences dangereuses sur le plan de la santé publique et de la préservation de l'environnement. C'est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, de favoriser une politique ambitieuse et cohérente de développement du système ferroviaire,

en inscrivant la lutte contre le réchauffement climatique comme cadre des décisions à prendre concernant l'avenir du rail français. En France, le secteur des transports est le principal émetteur de CO2 avec 39 % des émissions totales de gaz à effet de serre, augmentation de 10 % depuis 1990. Face à l'urgence écologique, le développement de modes de transport décarbonatés et verts est essentiel. Le train est dix fois moins émetteur de CO2 que la voiture, cinquante fois moins que l'avion.

lorsqu'elle considère que l'attribution directe est justifiée par les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau concernés, [ ...], et lorsqu'un tel contrat aurait pour effet d'améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux

Nous sommes satisfaits- une fois n'est pas coutume -que le Gouvernement ait proposé un amendement précisant ses intentions en la matière, en prévoyant la présence, au sein des organes de gouvernance du groupe public ferroviaire, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices, des associations d'usagers, ainsi que des représentants des personnels. Nous proposons simplement de préciser que cette représentation doit être significative.

Il s'agissait pour nous de prendre en compte la vision décentralisée du service de transport et de permettre aux salariés, comme aux usagers et aux élus, d'avoir une voix prépondérante pour que la politique de transport soit non pas guidée par des impératifs d'austérité budgétaire- cela a trop longtemps été le cas mais par les exigences de service public que porte l'ensemble des acteurs du quotidien du ferroviaire : les usagers, les personnels et les organisateurs de transport. Nous opposons aux politiques de concurrence des politiques de complémentarité, de meilleures réponses aux besoins de mobilité et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi- tel est l'objet de cet amendement -des objectifs de démocratisation des organes de décision des entreprises effectuant des missions de service public et détenues par la puissance publique. À nos yeux, tout l'intérêt de la maîtrise publique réside bien dans cette exigence d'un meilleur contrôle citoyen d'une entreprise financée par l'impôt et qui est l'outil de la Nation pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Aujourd'hui, trop de décisions ayant un impact direct sur le service public sont prises dans l'opacité par un nombre réduit de personnes, dont les intérêts sont identiques : réduire le coût de l'opérateur public.

À cet égard, la loi de 2014 était claire : les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement, et non fixés par décret ou ordonnance. Depuis des années, nous dénonçons le sous-investissement dans le réseau ferré. L'ouverture à la concurrence ne changera pas la donne ! Ce qu'il manque, c'est une politique volontariste d'investissements publics massifs. En effet, par nécessité d'améliorer la qualité du réseau, SNCF Réseau peut être amenée à réaliser des investissements, dont la finalité première ne serait pas la rentabilité- c'est bien la limite de la notion de règle d'or -, et à sélectionner des projets d'investissements selon des règles comptables obscures. La question n'est pas seulement celle de la trajectoire financière de SNCF Réseau, mais aussi celle des ressources nouvelles. Il est nécessaire d'acter de manière pérenne les priorités d'investissements ferroviaires de manière transparente et sur le long terme. C'est bien ce qui manque aujourd'hui en matière de politique industrielle. De nouvelles ressources sont envisageables, et nous avions fait de nombreuses propositions solliciter l'épargne populaire dans le cadre d'un « livret vert » dédié au financement des infrastructures de réseaux ou mettre à contribution les sociétés d'autoroute, dont les profits sont particulièrement insolents. La liste n'est pas exhaustive ! La priorité doit être donnée à la régénération du réseau ferroviaire et non à enserrer SNCF Réseau dans des contraintes budgétaires décidées loin des besoins des usagers et de nos territoires. Pis, nous ne pensons pas que le système ferroviaire peut s'autofinancer- c'est le propre de ce service public, structurant pour notre territoire. Madame la ministre, vous pouvez prendre le problème dans tous les sens, avoir un réseau de qualité avec un maillage territorial fin qui répond aux nouvelles exigences de mobilité coûte très cher, et le privé ne fera pas de miracle. C'est bien le désengagement de l'État qui est à l'origine de la dette

de l'infrastructure et l'exploitation des services de transport -est manifestement contraire au droit européen, qui, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, impose la séparation de ces activités. L'avis est donc

de légiférer par voie d'ordonnance pour déterminer les modalités de transformation du groupe public ferroviaire, qui est prévue à l'article 1 A. L'avis est donc défavorable.

... -vise à rétablir une précision : l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance prévue à l'article 1 permet de déterminer les conditions du transfert des biens, droits et obligations des établissements publics,

Par ailleurs, il est déjà clairement indiqué que l'habilitation doit permettre le transfert des biens, droits et obligations des établissements publics aux nouvelles sociétés anonymes.

un avis défavorable sur cet amendement. L'amendement n° 82 vise à préciser que la représentation des collectivités territoriales au sein de la gouvernance des entités du groupe public unifié devra être « significative

satisfaction ... Cet amendement vise à supprimer l'habilitation donnée au Gouvernement pour déterminer par voie d'ordonnance les règles de financement des investissements de SNCF Réseau.

« juste-à-temps » sur des parcours aléatoires et bien plus accidentogènes. Plutôt que de se demander s'il ne faudrait pas mettre un terme à l'emploi à vie qui découle du statut, il conviendrait de procéder à un renversement dialectique, en se demandant ce que l'expérience du statut des cheminots

On ne construit pas une économie développée digne de ce nom sur les ruines du droit du travail et l'extension permanente de la précarité et de la flexibilité, qui imposent au quotidien leur dure loi à des salariés en guerre les uns contre les autres. Le progrès économique de notre pays réside dans la qualité des statuts et des positions accordés aux salariés ; il découle de leur capacité à échanger, à coopérer et à partager leurs compétences et leurs qualifications pour le bien de la communauté que constitue l'entreprise et, dans le cas du transport ferroviaire, de la collectivité dans son ensemble. Mettre à mal le statut des cheminots- faut-il le dire ? -ne va rien régler des conditions de travail des chauffeurs routiers, des employés des compagnies d'autocar, ni, j'en suis sûr, des éventuels employés des compagnies ferroviaires qui viendraient concurrencer la SNCF. Le recul des droits des uns ne s'est jamais traduit, depuis la première réforme des retraites version Balladur, par l'avancée des droits des autres, car cette course au moins-disant social se paie toujours en fin de compte. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé dans la téléphonie mobile.

Pourquoi le Gouvernement a-t-il prévu au troisième alinéa de cet article le retour à l'État de tout ou partie des biens des EPIC ? N'y a-t-il pas un risque de voir SNCF Réseau dépossédée d'une partie de ses biens et qu'elle ne soit plus affectataire unique des infrastructures ferroviaires ?

Le scrutin est ouvert.

un droit de regard et d'intervention sur la mise en oeuvre de la politique ferroviaire, d'une part, en veillant particulièrement au contenu des contrats-cadres signés entre l'État et l'entreprise nationale SNCF et, d'autre part, en leur conférant un pouvoir d'avis sur ces projets de contrat et d'actualisation d'actualisation de ces mêmes contrats. Nous souhaitons ainsi nous assurer que ces contrats intègrent bien les attentes des pouvoirs publics, permettent le développement du service public et apportent des réponses effectives aux besoins en transport des usagers et des territoires. Qui mieux que la représentation nationale peut garantir cette prise en compte ? Actuellement, le projet de contrat-cadre n'est transmis qu'à l'ARAFER, ce qui nous semble extrêmement limité et insuffisant. Cette exigence semble rendue d'autant plus impérieuse par le changement de statut des entreprises publiques constituant le groupe public ferroviaire. Il importe que les organes démocratiques que sont le Parlement et le CESE soient associés étroitement à la préparation du futur contrat-cadre et de son actualisation, qui aura lieu en 2020. Celle-ci devra nécessairement prendre en considération les changements de mission du groupe ferroviaire. C'est un élément de transparence et de démocratie, sur lequel, je l'espère, nous arriverons à nous mettre d'accord.

de répondre comme elle le souhaite à cette transmission, notamment en organisant un débat ou une communication sur le sujet. Il ne me semble donc pas utile de prévoir un avis du Parlement. En conséquence, la commission

: La parole est à M. Alain Fouché. La réforme ferroviaire prévoit d'introduire SNCF Mobilités dans le champ de la concurrence. Dans cette optique, SNCF Mobilités ne devrait plus bénéficier de prérogatives qui pourraient constituer, dans cette nouvelle configuration, un avantage anticoncurrentiel par rapport aux autres compagnies. Il convient donc de supprimer ces prérogatives de gestion domaniale laissées à SNCF Mobilités, en modifiant le code des transports. Ces facilités doivent être réservées à l'EPIC de tête SNCF et à Gares & Connexions. Conformément à l'article L. 2141-13 du code des transports, SNCF Mobilités est compétente pour assurer la gestion domaniale de certains biens immobiliers appartenant à l'État ou qui lui sont confiés par convention avec l'État ou l'EPIC SNCF. Ces dispositions facilitent l'accès à des terrains ou à des logements qui peuvent être nécessaires au bon développement des services ferroviaires. Cette activité, qui constitue une activité commerciale, produit des revenus au profit de SNCF Mobilités. Dès lors, afin de garantir une concurrence équitable entre toutes les entreprises ferroviaires, il nous semble nécessaire d'inscrire dans le code des transports les principes résultant des règles de la comptabilité publique, qui imposent à tout opérateur en ou bénéficiant d'une position dominante d'établir des règles strictes de séparation comptable. En d'autres termes, il convient de garantir une stricte séparation entre les flux financiers issus de la gestion domaniale et ceux qui sont affectés à l'exploitation d'un service de transport. La deuxième partie de l'amendement vise à garantir que les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités et nécessaires à la poursuite des missions de transport doivent pouvoir être cédés

Cet amendement serait difficile à mettre en oeuvre s'il était adopté. Il tend à prévoir que les revenus que tire SNCF Mobilités de la gestion de ses biens immobiliers figurent dans des comptes distincts de ceux qui sont affectés à son activité de transport. La transformation de SNCF Mobilités en société anonyme nécessitera de revoir le régime des biens immobiliers qui lui sont affectés, en particulier des biens relevant du domaine public, qui pourront, le cas échéant, être transférés à l'État.

Sachez que l'affectation et le régime des biens au sein des différentes entités du groupe SNCF respecteront bien évidemment les règles en matière de droit de la concurrence. De ce point de vue, il faudra prévoir un traitement différent

afin de permettre non pas la recapitalisation de Fret SNCF, fusil à un coup dont l'objectif est de faire passer la filialisation-privatisation, mais bien le financement pérenne par l'État. Les institutions européennes bougent et évoluent en ce sens, comme en témoigne l'exemple italien. Il ne s'agit donc pas d'un simple amendement déclaratoire, mais bien d'un amendement aux conséquences précisées et directes : la possibilité pour l'État français de subventionner cette activité. Nous ne comprenons pas l'acharnement du Gouvernement et de la majorité sénatoriale à refuser de traiter cette question, reportant les enjeux sur d'autres sujets. La réalité est simple : la concurrence que vous imposez n'est pas compatible avec les enjeux environnementaux que nous défendons. Nous sommes en train de rater le coche, comme le prouve l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. Pourtant, l'enjeu est de taille. Selon plusieurs rapports, le volume de marchandises à transporter devrait être multiplié par trois au cours des quinze prochaines années. On assistera donc, globalement, à une explosion du transport de marchandises. Or, aujourd'hui, le fret ferroviaire ne représente que 10 % de ce trafic, alors que l'on avait fixé un objectif général de 25 %. Nous avons un boulevard. Il existe des besoins immenses d'investissement dans cette activité pour provoquer son essor : la remise à niveau des triages, des machines, des trains, des efforts concernant les infrastructures, mais également l'offre pour la développer. Permettre son subventionnement par l'État n'est donc pas une solution à rejeter d'un revers de main.

Cela passe aussi par des choix d'investissement que nous aurons à faire, notamment dans la continuité des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. Il s'agit d'avoir des sillons de qualité, une politique de péage adaptée et de promouvoir une politique d'aide au transport combiné. C'est l'ensemble de ces éléments qui constitue le plan de relance du fret ferroviaire que je présenterai prochainement. Je voudrais redire que le mouvement social actuel met en grande difficulté notre fret ferroviaire et les entreprises qui en dépendent. Tout à fait ! Je pense que la situation actuelle ne contribue pas à donner confiance dans le fret ferroviaire, et donc dans sa relance.

Le scrutin est ouvert.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

dans la politique de reconstruction nécessaire du fret ferroviaire. De toute façon, elle sera indispensable, mais nous espérons qu'elle sera mise en oeuvre avant que la catastrophe climatique et environnementale par l'envahissement des camions n'ait causé trop de ravages sur les routes de France et d'Europe.

Il n'en demeure pas moins que je suis particulièrement attentive aux changements apportés sur ces sites, qui ont besoin d'être remis en état, tout comme le réseau ferré principal.

objet est simple : créer de nouvelles ressources afin de pérenniser les financements du système ferroviaire à la fois pour le désendetter et pour renforcer l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Créée en 2004, l'AFITF a très vite été vidée de sa substance et des moyens qui lui étaient alloués, notamment avec la privatisation des autoroutes- nous en avons déjà parlé dans cet hémicycle -, à tel point que la Cour des comptes estime aujourd'hui qu'il s'agit d'une coquille vide. Autant dire que cette agence n'a pas les moyens de ses ambitions, lesquelles, d'ailleurs, sont réduites à très peu. En effet, il manquerait dans son budget, pour les cinq ans à venir, quelque 10 milliards d'euros. La mission d'intérêt général du transport ferroviaire est d'assurer un maillage suffisant du territoire national et de proposer un mode de transport non émetteur de gaz à effet de serre. toutes et tous d'accord ici. C'est pourquoi il est impératif de dégager des ressources à même de financer des investissements de rénovation, ainsi que de nouveaux projets. Pour ce faire, en vertu du principe pollueur-payeur », nous proposons que la route finance le rail, d'où la renationalisation des autoroutes. La manne financière que constitue cette rente s'élève à près de 2 milliards d'euros et serait beaucoup plus utile dans les caisses de SNCF Réseau que dans les poches des actionnaires d'Eiffage ou de Vinci. Dans la même logique, nous proposons la mise en oeuvre d'une écotaxe poids lourds, qui sera à même de lever 1 milliard d'euros supplémentaires et qui aura également un effet incitatif pour favoriser le fret ferroviaire, que vous appelez de vos voeux, madame la ministre, si j'ai bien compris. L'adoption de cet amendement pérenniserait les financements du système ferroviaire tout en renforçant l'effort de transition écologique dans le secteur du transport. La question du financement des investissements nécessaires à la remise en état du réseau ferré comme à son développement à venir est évidemment directement posée par le présent projet de loi. On aura observé que le changement de statut de la SNCF prévu par le texte présente, de ce point de vue, un risque. En effet, même si elle donne quelques poussées d'urticaire aux instances européennes, l'actuelle forme juridique de la SNCF, à savoir celle d'un EPIC, lui donne un accès de grande qualité aux marchés financiers, par la combinaison du caractère de long terme de l'investissement ferroviaire et du statut d'EPIC. De fait, l'EPIC SNCF bénéficie d'une « garantie implicite et illimitée de l'État », ce qui lui permet à la fois de négocier des emprunts à taux et à conditions privilégiés et d'être prémuni contre tout défaut de paiement. Pascal Savoldelli en a déjà parlé, mais je préfère rappeler aux adeptes de la transformation de la SNCF en société anonyme à capitaux d'État que l'abandon du statut d'EPIC risque fort de conduire à la « banalisation » des financements accordés à l'entreprise, donc à une remontée des taux d'intérêt grevant sa dette. vrai que, bien qu'activement gérée, la dette de la SNCF a un aspect « boule de neige », qui se traduit par une forme de fuite en avant, les intérêts de la dette amortie devenant le capital de la dette inscrite au bilan. Ajoutons qu'un ajustement comptable à 12 milliards d'euros a ruiné les fonds propres du groupe Il est donc temps de se demander s'il n'y aurait pas lieu de créer, comme nous le proposons, un livret d'épargne défiscalisée, sur le modèle du livret A ou du LDD, pour financer les investissements ferroviaires et, de manière plus générale, les investissements nécessaires à l'atteinte de nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques.

De son côté, le Gouvernement a annoncé qu'il présenterait prochainement un plan de relance du fret ferroviaire. Pour ce qui nous concerne, nous considérons que mener un bilan de l'ouverture du fret à la concurrence engagée en 2006 constitue un préalable. Le soutien au fret ferroviaire est est indispensable du fait des externalités positives qu'il représente, en termes de réduction des émissions de dioxyde de carbone. Cette activité doit demeurer sous maîtrise entièrement publique, car elle constitue un levier fondamental de la transition énergétique. énergétique. Il paraît donc aujourd'hui prématuré de filialiser cette activité, cette filialisation pouvant constituer une étape vers son externalisation et sa privatisation. Par ailleurs, dans son référé du 3 juillet 2017 sur la situation du transport de marchandises par le groupe SNCF Mobilités, la Cour des comptes a souligné que, à défaut d'un dispositif financier permettant de prendre en compte les externalités négatives de la route, qui aurait pu durablement inciter les chargeurs à se reporter sur le transport ferroviaire, l'État devrait pouvoir afficher une stratégie de long terme de soutien au fret ferroviaire, qu'il s'agisse de la pérennité des aides financières aux opérateurs de combiné (aide à la pince) ou du maintien de la compensation aux péages fret, permettant de maintenir l'attractivité de ce mode de transport face à l'aptitude très forte de la route à comprimer ses coûts ». Or l'actualité européenne nous rattrape.

Le rail devrait donc pouvoir bénéficier à un horizon proche de nouvelles ressources financières, raison pour laquelle le fret ferroviaire en tant que levier de la transition énergétique doit rester public et intégré dans le groupe public SNCF. Pour toutes ces raisons, nous estimons que le plan de relance du fret ferroviaire doit être conçu dans la perspective de ces nouvelles ressources financières. Nous demandons donc que le Gouvernement remette au Parlement

Vous connaissez mon allergie à cette multiplication des demandes de rapport, qui, il faut bien le dire, servent souvent à pallier l'absence de mesures véritables et qui mobilisent des effectifs importants dans les ministères, sans être généralement suivis d'effets concrets.

du développement des infrastructures et des financements correspondants, l'objectif étant bien de disposer désormais d'une vision pluriannuelle, avec une programmation équilibrée

8, cette directive dispose : « Les États membres développent l'infrastructure ferroviaire nationale en tenant compte, le cas échéant, des besoins généraux de l'Union, y compris celui de coopérer avec les pays tiers voisins. Ils publient, à cette fin, au plus tard le 16 décembre 2014, après consultation des parties intéressées, une stratégie indicative de développement de l'infrastructure ferroviaire visant à répondre aux futurs besoins de mobilité en termes d'entretien, de renouvellement et de développement de l'infrastructure et reposant sur un financement durable du système ferroviaire. Cette stratégie couvre une période d'au moins cinq ans et est reconductible. « Dans le respect des articles 93, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres peuvent en outre accorder au gestionnaire de l'infrastructure un financement compatible avec ses fonctions visées à l'article 3, point 2, la dimension de l'infrastructure et les besoins financiers, notamment pour couvrir des investissements nouveaux. Les États membres peuvent décider de financer ces investissements par des moyens autres que le financement direct par l'État. En tout état de cause, les États membres se conforment aux exigences visées au paragraphe 4 du présent article. point 1, entre autres conclusions, que la Banque centrale européenne a un rôle particulier à jouer dans le financement des infrastructures ferroviaires de l'ensemble de l'Union européenne, notamment pour la reprise de la dette. Quant au point 2, il nous montre que notre proposition de livret d'épargne est cohérente et correspond aux possibilités de financement retenues.

le développement touristique, et j'en passe. Elle peut demain, si on le décide, participer au financement de la transition énergétique et écologique, singulièrement par le renouvellement et le développement de notre réseau ferroviaire.

vote. Comme j'ai tenté de l'expliquer, sans un moteur financier particulier pour discriminer positivement le fret ferroviaire, on continuera à produire de beaux discours et à sortir je ne parle même pas des rapports, monsieur le rapporteur. La situation du fret démontre notre impuissance collective, alors qu'il y a unanimité politique sur cette question. D'ailleurs, dans le texte, on ne trouve pas de dispositif qui permette de résoudre l'inégalité de traitement que subit le transport ferroviaire, pourtant

à la transition énergétique et de mieux organiser le flux routier en traitant la question du fret, qui apparaît trop peu ici. Quand il est moins cher de traverser le pays en avion ou en bus qu'en train, il faut s'interroger sur ce besoin d'un dispositif adapté. Il faut aussi sortir d'une logique malthusienne dans le transport ferroviaire, qui est une industrie de réseau. Plus on fait rouler de trains sur les voies, plus on baisse les coûts unitaires, en travaillant sur le coût marginal. C'est une démonstration qu'a su faire la Suisse en faisant rouler des trains de fret la nuit,

du fret routier. Si l'on veut améliorer la qualité de l'air, il faudra bien évoquer ce sujet un jour, mais dans une vision territoriale et apaisée. En tout état de cause, je ne crois pas que c'est au détour d'un amendement que nous pourrons envisager un dispositif respectueux des territoires. ailleurs, je m'inscris en faux contre un rapprochement hâtif des dates : l'ouverture à la concurrence du fret n'a pas eu les mêmes conséquences partout. En Allemagne, avec les mêmes dates, elle s'est traduite par une augmentation du fret ferroviaire. Il faut donc chercher ailleurs

pour tenter de résoudre un problème de péréquation, qui, en vérité, découle de la logique dans laquelle la loi nous entraîne et risque de mettre en très grande difficulté les lignes dites « déficitaires

nous sommes de grands défenseurs des territoires. Il faut faire en sorte que l'ensemble des TGV irriguent le territoire avec des dessertes directes, sans correspondance.

pour un certain nombre de dessertes, auxquelles le Gouvernement est attaché. C'est bien parce que nous sommes attachés à la desserte de nos territoires par le TGV et que, par ailleurs, nous pensons qu'une ouverture à la concurrence, sous forme de franchises, aurait été beaucoup plus violente pour la SNCF que nous avons proposé ce système, qui conduit à procéder à une péréquation, celle qui existe actuellement pour les comptes de l'activité TGV, au travers des péages. Dans le même temps,

en accord avec l'ARAFER, qui souscrit tout à fait à l'intérêt de ce dispositif, le Gouvernement souhaite utiliser la péréquation au sein des péages afin d'assurer le maintien

De nombreuses collectivités territoriales situées en deçà ou au-delà du tracé des lignes à grande vitesse ont participé à leur financement, en échange d'une desserte de leur gare par des trains à grande vitesse

du tracé de lignes à grande vitesse à avoir contribué à leur financement, afin de garantir la desserte de leur gare par des trains à grande vitesse et, par là même, d'éviter les potentielles ruptures de charge dont pourraient souffrir leurs usagers. amendement entend sécuriser lesdites dessertes, en précisant que le calcul des redevances d'infrastructure perçues par SNCF Réseau devra prendre en compte la nécessité pour l'État de respecter les engagements pris lors de la construction des lignes à grande vitesse à l'égard des collectivités territoriales concernées.

Allez

Alors que le présent article reprend uniquement l'idée d'une modulation en fonction de l'intérêt des lignes en matière d'aménagement du territoire, nous souhaitons élargir les critères de définition du niveau de péage.

Ainsi, l'utilisation de matériel de traction diesel par certains opérateurs sur des lignes électrifiées pourrait être pénalisée en augmentant les péages, tandis que celle de rames de TGV à deux étages, moins consommatrices de sillons, pourrait être encouragée par une minoration de ces

Nous pensons que la possibilité de modulation pour raisons écologiques s'avère indispensable pour optimiser la gestion des flux et l'utilisation des réseaux. Quel est l'avis de la

Dès lors que la problématique des dessertes visées par les auteurs de ces amendements est d'ordre tarifaire, ces amendements sont pleinement satisfaits par le critère du maintien

un tel ajout n'aura aucune portée. Il ne revient pas à l'outil tarifaire de résoudre des problèmes plus généraux entre des collectivités territoriales et l'État quant au respect d'engagements, dont la forme n'est d'ailleurs pas précisée. En tout état de cause, cet ajout sera sans doute inapplicable pour le gestionnaire d'infrastructure et l'autorité de régulation, car je ne vois pas comment ils pourront se référer à des éléments objectifs et précis. Cela ne remet pas en cause le bien-fondé de ces amendements, qui témoignent de l'inquiétude des élus locaux dans certains territoires quant à la cohérence dans le temps des décisions de l'État sur les lignes à grande vitesse. Nous comprenons parfaitement le message politique

Nous ne pensons pas que le législateur, le Sénat, ait à introduire de telles distinctions dans la loi. Que penseront les élus de tous les territoires dont la desserte n'était pas prévue une LGV ? Ils pourront avoir l'impression légitime d'être oubliés par le législateur. Si nous visons des situations particulières sans être exhaustifs, nous allons susciter de nouvelles demandes, car certains élus ou concitoyens auront légitimement l'impression d'avoir été oubliés ou lésés. Pourquoi ne pas viser les dessertes situées en zone de montagne ou encore en zone de revitalisation rurale ? Privilégions la concision dans la loi,

pris notamment dans le cadre des conventions de financement d'un certain nombre de lignes à grande vitesse soient respectés. Tel est d'ailleurs le sens de la péréquation qui est proposée.

doit permettre l'équilibre de la plupart des dessertes. Le cas échéant, tel est bien le sens des compléments qui ont été apportés par la commission, il faudra prévoir

sous-entend que certaines d'entre elles ne seront pas en équilibre financier. Selon le chiffre qui avait été donné lors de votre audition par M. Maurey,

il faut un contrôle démocratique de cette question, ce que nous proposerons par une programmation de la notion de desserte d'intérêt national, et un vrai débat sur cette question. J'ai bien compris la

le maintien des dessertes. Si les collectivités territoriales ont mis la main à la poche, c'était pour obtenir une garantie. Élu de Bretagne, je me souviens des discussions- je me tourne vers mon collègue Louis-Jean de Nicolaÿ -sur le maintien de la desserte du Mans.

au moment du montage du dossier. l'ouverture à la concurrence ne va pas la conduire à déchirer cet engagement. Elle ne pourrait en être déliée que si elle démontrait que l'évolution de la concurrence, par exemple l'arrivée d'un opérateur qui écrémerait le marché sur cette ligne, la met dans l'impossibilité de respecter ses engagements.